La séance est reprise. J’informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels est parvenue à l’adoption d’un texte commun.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

amendement vise à défendre un principe simple, mais fondamental, en instaurant une représentation plus complète et plus juste au sein du comité d’attribution. Il s’agit de permettre aux élus locaux, aux représentants de l’État et aux parlementaires de jouer un rôle plus actif et décisif dans ce processus crucial. Cette modification incarne la volonté de donner la possibilité à ceux qui connaissent le mieux les territoires ultramarins de partager avec l’État les priorités de ces territoires. C’est une question non seulement d’équité ou de représentativité, mais aussi de responsabilité envers les communautés locales, qui sont en symbiose avec les besoins et les aspirations de ceux qui habitent et travaillent sur ces territoires. la mesure où il sera composé de représentants de l’État, des collectivités – ou de la collectivité – et des parlementaires, s’inscrit parfaitement dans la logique de l’expérimentation proposée dans l’amendement de Mme Conconne. Il s’agit là d’une synergie vertueuse qui vise à tester une approche innovante et inclusive pour stimuler le développement des territoires ultramarins, dont je rappelle qu’il doit être en faveur de nos concitoyens. En conclusion, mes chers collègues, ce sous amendement n’est pas simplement une réforme administrative, il représente un engagement en matière de justice, d’équité

Le bénéfice de cet article doit être limité aux personnes dont les ressources ne dépassent pas la moitié du plafond de la sécurité sociale. Je vous fais pleinement confiance sur ce sujet. Vous et vos collègues savez faire et avez l’habitude de conditionner des aides.

Le premier écueil est constitutionnel. En effet, comment cibler sans exclure ni catégoriser, tout en restant conforme aux principes républicains ? Ce n’est pas si simple, surtout lorsque l’on se rappelle la nomination de délégués interministériels à l’égalité des chances des Français d’outre mer. Le deuxième point de vigilance porte sur les attentes des populations, telles que les expriment leurs représentants. En effet, l’éloignement géographique est un obstacle matériel à un projet de retour, eu égard au coût que cela peut représenter. Enfin, on peut s’inquiéter de ce que le dispositif encourage le retour dans des territoires où le taux de chômage est préoccupant.

Naminzo. Il s’agit d’un amendement de repli. Alors que le droit à une continuité territoriale cohérente et complète pour tous les ressortissants des territoires d’outre mer semble encore trop difficile à garantir,

tenir compte des intérêts matériels et moraux.

pour présenter l’amendement n° II 1183 rectifié. Cet amendement vise à modifier les contours du passeport pour la mobilité en stage professionnel, afin de mieux accompagner les élèves et les étudiants ultramarins devant effectuer, dans le cadre de leur cursus, un stage, une alternance ou un déplacement hors de leur collectivité d’origine. Actuellement, l’aide ne peut être attribuée qu’aux étudiants inscrits jusqu’au niveau master, ce qui exclut de fait les étudiants de certaines filières. Je pense notamment aux étudiants en médecine qui disposent souvent de faibles revenus et qui doivent effectuer de nombreux stages de spécialisation. Cet amendement vise donc à élargir le public cible du passeport, afin de permettre à tout étudiant inscrit dans l’enseignement supérieur et suivant une formation initiale de bénéficier de la prise en charge de son titre de transport. Il tend également à étendre le bénéfice de cette aide aux élèves et étudiants ultramarins en alternance, pour tenir compte du développement de l’apprentissage dans nos territoires et dans l’Hexagone. Afin de couvrir tout le spectre des formations à distance, cet amendement a enfin pour objet de permettre la prise en charge des mobilités qu’induisent les études à distance pour les examens en soutenance hors de la collectivité de résidence des étudiants.

que les envois entre particuliers depuis l’Hexagone : ce dispositif est donc aussi incomplet qu’inefficace. Or le désenclavement de nos territoires d’outre mer appelle des mesures fortes. Du fait de leurs études ou de mutations dans la fonction publique d’État, les Réunionnais sont toujours contraints à se rendre dans l’Hexagone. Dès lors,

s’agit donc d’un enjeu significatif présentant de multiples facettes. Il y a urgence à agir, d’autant que les ménages ultramarins ont un niveau de vie bien inférieur à celui des habitants de l’Hexagone. L’accès au logement en outre mer est d’autant plus inabordable que 80 % des Ultramarins sont éligibles au logement social,

Il a été adopté à l’Assemblée nationale, mais n’a pas été retenu après l’utilisation du 49.3 par le Gouvernement. Nous le proposons de nouveau aujourd’hui, afin de lancer le plus rapidement possible un grand plan d’investissement pour les infrastructures de distribution d’eau potable dans lesdits territoires.

En dehors des restrictions, l’accès à l’eau potable n’existe toujours pas ou n’est que partiel pour une part encore très importante des populations ultramarines. En Guyane, près de 20 % de la population n’a pas du tout accès à l’eau potable à son domicile

pour garantir l’accès à l’eau potable pour tous et pour toutes dans les territoires ultramarins. C’est pourquoi nous proposons ce plan d’urgence sur l’eau dans les territoires d’outre mer. Il vise à financer prioritairement le renouvellement et l’amélioration des réseaux de distribution d’eau pour mettre fin aux fuites et pour adapter les territoires aux aléas climatiques. Il vise également à financer la mise en place de systèmes d’assainissement efficients dans tous les territoires et l’établissement de plans de dépollution et de prévention des pollutions pour protéger la ressource.

je formalise simplement l’amendement de la manière suivante : abonder à hauteur de 50 millions d’euros d’autorisations d’engagement et de crédits de paiement l’action n° 08 « Fonds exceptionnel d’investissement » du programme 123 « Conditions de vie outre mer

des départements et régions d’outre mer. De nombreuses mesures ont été mises en place ces dernières années pour renforcer la capacité de certains territoires, notamment Mayotte, la Martinique et la Guadeloupe, à gérer la ressource au travers d’un appui aux syndicats mixtes de gestion des eaux et d’investissements dans les infrastructures. En complément de ces mesures prises en direction des collectivités, il importe de travailler sur les usages de l’eau. De ce point de vue, les entreprises sont des usagers de premier rang. Le présent amendement vise à les soutenir dans l’optimisation de leurs processus industriels en matière de consommation de Le dispositif proposé pourrait être confié à l’Office français de la biodiversité et prendrait la forme d’un appel à projets simplifié à destination des entreprises souhaitant moderniser

PEC est à la fois un levier d’insertion professionnelle pour les personnes éloignées de l’emploi et, de fait, un élément indispensable au bon fonctionnement des collectivités. Quel

pour défendre un amendement vital visant à accroître les crédits alloués aux contrats de convergence et de transformation (CCT) ainsi qu’aux contrats de développement (CDEV) du programme « Conditions de vie outre mer vie outre mer ». Bien plus que de simples documents administratifs, ces contrats sont une opportunité pour nos territoires ultramarins de s’engager dans des projets structurants, de répondre aux enjeux écologiques et environnementaux cruciaux et de façonner un avenir durable pour nos communautés.

Je suggère également de réduire dans les mêmes proportions les moyens de l’action n° 02 du programme 138 « Emploi outre mer ». Cette réaffectation budgétaire n’est pas simplement un déplacement de fonds d’une catégorie à une autre, elle est un investissement ciblé qui garantira le développement durable et la prospérité de nos territoires ultramarins. En renforçant les CCT et les CDEV, nous donnons aux collectivités locales les moyens nécessaires pour bâtir un avenir meilleur, où développements écologique et économique vont de pair. Je vous appelle donc à soutenir cet amendement crucial en investissant dans nos territoires d’outre mer. Nous semons aujourd’hui les graines d’une croissance durable et inclusive

qui correspond à un montant de 5 millions d’euros d’aide au fret qui aurait dû être octroyé à la filière, mais que les acteurs locaux ont dû assumer eux mêmes, met en péril l’autonomie alimentaire de l’île, alors qu’elle dépend déjà beaucoup des importations. Les éleveurs réunionnais, tout comme l’ensemble des filières, nous rappellent la nécessité de contenir les prix en soutenant la productivité locale et de participer plus largement à la lutte contre le coût de la vie. Un soutien à la production locale de fruits et de légumes de 10 millions d’euros a été mis en place pour compenser les surcoûts liés à la guerre en Ukraine, mais son caractère conditionnel se révèle trop contraignant.

et l’absence de trésorerie pèse sur la production locale. Dès lors, il faut revoir le conditionnement de ce soutien et – surtout – l’ouvrir au plus grand nombre afin de venir vraiment aux agriculteurs ultramarins. C’est ce que nous proposons. La moitié des fruits et légumes consommés à La Réunion sont issus de la production locale : c’est un bon résultat comparé à d’autres territoires, mais – comme je l’ai souligné – la situation est fragile. Il faut s’assurer qu’elle ne se dégrade pas et aller plus loin pour que l’autonomie alimentaire soit une réalité outre mer. Il s’agit, au travers de cet amendement, de reconduire le dispositif de soutien à la production locale pour 2024.

En 2022, l’AFD a accordé 906 millions d’euros de prêts au secteur public ultramarin, dont 365 millions d’euros concernaient des prêts bonifiés par l’État. Les bonifications de prêt de l’AFD permettent donc aux collectivités et aux établissements publics ultramarins de jouir d’un accès aux financements à des taux très avantageux pour leurs projets de développement durable dans les territoires qui en ont le plus besoin. Nous constatons que 1 euro de bonification permet d’engendrer 10,50 euros de financements. Cependant, dans un contexte de remontée des taux d’intérêt, les collectivités locales rencontrent des difficultés pour financer leurs projets structurants. Cette dotation supplémentaire aidera les acteurs publics des outre mer à poursuivre leurs engagements en faveur des projets essentiels pour leurs territoires, en particulier pour les enjeux écologiques et environnementaux.

Ainsi, l’enveloppe de bonifications allouée à l’AFD pour 2024 serait portée à 44,185 millions d’euros, contre 34,185 millions d’euros notifiés en loi de finances initiale pour 2023. Quel

Cour des comptes de juin 2022,, 84 % de la population de Mayotte vit sous le seuil de pauvreté. Alors que le territoire de Mayotte est confronté à une situation d’extrême pauvreté, les dispositifs de lutte contre la précarité alimentaire constituent souvent un filet de sécurité pour les publics les plus précaires. Cette logique a eu tendance à s’accroître avec la crise sanitaire et ses conséquences sociales induites. C’est pourquoi, au travers de cet amendement, nous proposons d’augmenter de 5 millions d’euros les crédits du programme « Conditions de vie outre mer au profit d’un chèque alimentaire d’urgence pour Mayotte. Ce chèque alimentaire est une mesure d’urgence, mais aussi une mesure sanitaire et un impératif social et économique puisque la nourriture, à Mayotte, coûte bien plus cher que dans l’Hexagone. L’objectif est de pouvoir réduire le poids de l’insécurité alimentaire sur le territoire, d’augmenter les réponses à destination de l’ensemble de la population en faveur d’une alimentation de qualité et en quantité suffisante. En attendant la mise en place de mesures structurelles de long terme que nous appelons de nos vœux, nous proposons la création

Dès lors, conformément à l’organisation de nos travaux décidée par la conférence des présidents et en accord avec la commission des finances, la suite de l’examen de cette mission est reportée à demain, vendredi 8 décembre, en dernier point de l’ordre du jour, à l’issue de l’examen de la mission « Agriculture, alimentation,

il me revient de vous présenter, en quelques minutes, la position de la commission des finances sur les trois missions et le compte d’affectation spéciale qui couvrent le périmètre de Bercy. La commission vous proposera d’adopter l’ensemble de ces crédits, sous réserve de leurs modifications par quelques amendements. Je commencerai par la mission « Gestion des finances publiques Elle porte les crédits d’administrations cruciales pour la gestion des dépenses et des recettes de l’État ainsi que pour nos concitoyens, puisqu’il s’agit de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de la direction générale des douanes et des droits indirects Pour vous donner l’appréciation de la commission sur les crédits demandés sur cette mission, je dirai qu’il s’agit d’un budget de reconduction, mais d’une reconduction à un niveau élevé. L’année 2023 avait en effet interrompu dix ans de baisse par une hausse inédite des crédits. L’année 2024 s’inscrit dans cette dynamique, avec quasiment 11 milliards d’euros. On est donc loin, monsieur le ministre, du retour à une trajectoire de stabilisation annoncée l’an dernier. Bien sûr, certaines évolutions sont tout à fait positives. Je pense, par exemple, à l’achat de matériels de détection pour la douane, à la sécurisation des conditions d’exercice des contrôleurs fiscaux, au renforcement du renseignement douanier ou encore à l’octroi de moyens supplémentaires pour Tracfin afin de lutter contre les flux de financement illicites. Sur le temps long, toutefois, c’est à dire depuis dix ans, il convient de noter que les crédits n’ont augmenté que de 1,16 %. De fait, la mission « Gestion des finances publiques » a souvent été la seule à s’inscrire dans une logique de rationalisation des dépenses. C’est un effort qu’il convient de De même, sur ces deux dernières années, les crédits ont augmenté moins vite que l’inflation. Je dirai quelques mots à présent sur la mission « Crédits non répartis ». La provision relative aux rémunérations publiques fait l’objet cette année d’une ouverture de crédits à hauteur de 285,5 millions d’euros. Ils seront essentiellement consacrés au volet « Prévoyance » de la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics de l’État. Je regrette, monsieur le ministre, de constater chaque année la dégradation de la qualité des informations transmises par le Gouvernement sur les mesures financées par cette dotation. qui concerne la dotation pour dépenses accidentelles et imprévisibles, son examen annuel ne peut que provoquer une certaine lassitude. Le Gouvernement a pris l’habitude, depuis la crise sanitaire, de proposer des ouvertures excessives sur ce programme.

Les montants demandés demeurent en effet très largement supérieurs aux montants exécutés ces dernières années. La commission présentera donc, dans un souci de « sincérisation » budgétaire, un amendement de minoration des crédits de cette dotation. Je passe maintenant à la mission « Transformation et fonction publiques », sur laquelle je souhaiterais partager deux observations. En premier lieu, je voudrais souligner l’augmentation de près de 50 % des autorisations d’engagement prévues en 2024, qui atteindraient le niveau inédit de 1,2 milliard d’euros. Les crédits de paiement se stabiliseraient à un niveau élevé de 1,1 milliard d’euros. M. le ministre nous dira peut être que c’est le signe que la mission présente enfin la montée en charge tant attendue. Pour une mission créée en 2018 et qui avait vocation à s’éteindre en 2022, on n’aurait finalement que deux à trois ans de retard… J’en veux pour exemple les cités administratives : leur rénovation devait s’achever en 2022, mais l’enveloppe de crédits la plus importante serait En second lieu, je note que la mission continue d’être affectée par des défauts structurels, en dépit de quelques progrès. J’ai parlé du programme 348 en évoquant les cités administratives. J’ajouterai juste que le retard constaté s’est mécaniquement accompagné d’une augmentation des coûts sous l’effet de l’inflation. neuf chantiers prévus en 2018, trois ont été abandonnés et seules cinq cités ont été livrées à ce jour. De même, les crédits consacrés au programme « Transformation publique » continuent de connaître une sous consommation récurrente,

pourquoi la commission présentera un amendement de sincérisation budgétaire des crédits de la mission. Enfin, je conclurai brièvement sur le compte d’affectation spéciale (CAS) « Gestion du patrimoine immobilier de l’État les crédits s’élèveraient à 340 millions d’euros en 2024. La diminution de près de 30 % par rapport à 2023 s’explique principalement par l’évolution des recettes, marquée par une chute de 40 % des produits de cession. Ainsi, au regard de Ainsi, au regard de la valeur totale du patrimoine de l’État, estimé à 73 milliards d’euros, le CAS constitue actuellement un outil marginal. La parole

En premier lieu, nous notons que la progression de 1,5 % des crédits de la mission « Régimes sociaux et de retraite » est directement liée à la dynamique inflationniste et à la revalorisation des pensions qu’elle induit, à hauteur de 5,3 % au 1 janvier 2024. Les subventions d’équilibre versées aux régimes de la SNCF et de la RATP représentent encore, malgré la fermeture respective de ces régimes en 2020 et en 2023, 70 % des crédits de la mission. Les deux tiers des charges de pensions de ces régimes seront ainsi financés par le contribuable en 2024. La commission se félicite que la mise en œuvre de la réforme des retraites permettra de faire contribuer davantage les affiliés des régimes spéciaux à leur financement.

un texte expurgé de l’amendement voté par le Sénat sur ma proposition, et qui tendait précisément à garantir la compensation intégrale, chaque année, de la charge induite pour le régime général. Concernant le compte d’affectation spéciale « Pensions », il est désormais certain que son solde cumulé deviendra déficitaire d’ici à 2026 et que le relèvement de la contribution employeur de l’État sera nécessaire pour assurer la continuité du versement des pensions des fonctionnaires. La commission considère que ce relèvement doit intervenir au plus vite et de manière progressive afin de lisser son effet sur les budgets des ministères. Il est regrettable que le Gouvernement n’ait pas pu ou voulu m’apporter les précisions demandées sur le calendrier de mise en œuvre et sur son ampleur.

La réforme devrait justement permettre de limiter le niveau du relèvement nécessaire de la contribution employeur de l’État en réduisant le déficit du régime de 300 millions d’euros en 2025 et de 1,2 milliard d’euros d’ici à 2035. En tout état de cause, compte tenu de la nécessité de permettre le versement sans interruption des pensions des assurés des régimes spéciaux et des fonctionnaires de l’État, la commission s’est déclarée, sous ces réserves,

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, les crédits du programme « Fonction publique », de la mission « Transformation et fonction publiques qui financent le volet interministériel de la politique de ressources humaines de l’État, sont, à périmètre constant, en légère augmentation par rapport à la loi de finances pour 2023, avec 275,8 millions d’euros en autorisations d’engagement.

insuffisamment rigoureux et en partie subjectifs. Je vous proposerai tout à l’heure deux amendements visant à préciser les indicateurs relatifs aux prestations d’action sociale et au recrutement dans la fonction publique. D’autre part, je ne peux que déplorer les conséquences de la suppression, en loi de finances initiale pour 2023, du rapport sur l’état de la fonction publique et des rémunérations, jusqu’alors annexé au projet de loi de finances.

la date de parution de ce rapport est très aléatoire : j’en veux pour preuve qu’il n’est toujours pas paru, alors que nous sommes le 7 décembre. Cette situation ne permet pas au Parlement d’exercer ses missions dans des conditions satisfaisantes. Je pense que vous en conviendrez. conviendrez. Sur le fond, ensuite, les modalités de financement de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale me semblent très préoccupantes. Vous le savez, la loi de finances pour 2023 a acté le désengagement financier de l’État à ce sujet.

Mais cette apparente stabilité ne doit pas nous tromper : dès 2024, la contribution versée par France Compétences diminuera, et nous ne disposons à l’heure actuelle d’aucune garantie concernant le montant qui sera versé par l’État au delà de 2025. À moyen terme, c’est bien l’équilibre du système de financement, donc le développement de l’apprentissage public, qui est menacé. À l’heure où l’apprentissage dans la fonction publique territoriale constitue une composante à part entière de la politique des ressources humaines des collectivités territoriales,

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, 2024 est une année particulière, puisqu’elle est la première année de pleine application de la réforme paramétrique des retraites de 2023, votée dans les conditions que nous avons tous à l’esprit au printemps dernier et entrée en vigueur à compter du 1 septembre 2023. Avant d’entrer dans le détail des crédits de la mission et du compte d’affectation spéciale,

sont très claires : si le recul de l’âge de départ doit permettre, à moyen terme, de limiter le flux des départs à la retraite, il ne suffira pas à compenser la hausse des dépenses de retraite, qui devrait induire, selon les projections du COR,

vers les régimes de retraite spéciaux des agents de la SNCF et de la RATP. Il convient de rappeler que la réforme paramétrique n’a pas d’effet significatif sur les dépenses des régimes de la SNCF et de la RATP, dès lors que le Gouvernement a prévu qu’elle n’entrerait pas en vigueur avant le 1 janvier 2025 pour ces deux régimes. La réforme de 2023 a néanmoins eu pour effet de fermer aux nouveaux entrants le régime de la RATP à compter du 1 septembre 2023. Depuis cette date, les nouveaux agents de la RATP sont affiliés au régime général. Cependant, la caisse de retraite de la RATP reste responsable du paiement et de la liquidation des cotisants qui étaient affiliés au régime avant sa fermeture, et la date d’extinction effective du régime devrait intervenir aux alentours de 2116. C’est dans ce contexte que le Gouvernement a engagé une remise en cause du schéma de financement actuel des régimes spéciaux, par l’article 15 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, considérée comme définitivement adopté en application de l’article 49.3 de la Constitution depuis ce lundi 4 décembre. Dans le schéma proposé, l’ensemble des régimes spéciaux fermés seront intégrés financièrement à la Cnav. Par conséquent, l’État ne versera plus de subvention d’équilibre annuelle pour ces régimes, mais affectera au régime général une fraction de TVA de TVA visant à compenser globalement les charges associées à ces compensations d’équilibre. Cette nouvelle architecture de financement aura pour conséquence de vider la mission « Régimes sociaux et de retraite » de 87 % de ses crédits. Elle soulève deux préoccupations majeures. Premièrement, l’architecture proposée réduit la lisibilité du financement par la solidarité nationale des régimes spéciaux. Deuxièmement, elle a pour effet de dessaisir le Parlement de sa mission de vote annuel et de contrôle sur ces subventions d’équilibre. Je me félicite cependant que le Gouvernement ait conservé, dans le texte définitif, l’amendement de la commission des affaires sociales du Sénat

se trouve dans une conjoncture particulièrement délicate, en raison de la hausse dynamique de ses dépenses, liée à l’indexation des pensions sur l’inflation, et de la hausse plus modérée de ses recettes. Le résultat de ces deux tendances est un déficit croissant du CAS « Pensions », qui atteindra 2,5 milliards d’euros en 2024 et qui est estimé à 4,6 milliards d’euros

Nous souhaitons de la lisibilité sur l’évolution des paramètres qui aura pour conséquence de réintégrer, à moyen terme, plus de 4 milliards d’euros dans les crédits des missions du budget général. Mes chers

récemment, le collectif Nos services publics dénonçait « le sentiment croissant d’urgence et de dégradation des services publics », qui « s’exprime essentiellement à travers un discours déplorant des services publics qui s’effondrent et Républicain sont très attachés aux services publics, qui sont un rempart contre les inégalités sociales. Ils sont notre patrimoine commun et le seul capital de ceux qui n’en ont pas. C’est pourquoi nous portons une attention particulière aux fonctionnaires, à ces hommes et ces femmes qui œuvrent tous les jours pour accueillir au mieux le public dans nos administrations locales, nationales, sociales, nos écoles, nos commissariats, nos agences des finances publiques. Au travers de ce débat budgétaire, c’est aussi notre vision du service public, de l’organisation de l’État et de la fonction publique

aux collectivités, en passant par les hôpitaux, toutes les catégories de la fonction publique sont malheureusement touchées. La stigmatisation des fonctionnaires – ils seraient trop nombreux, trop coûteux, trop revendicatifs, pas assez productifs…

d’abord du temps de travail. En 2019, la loi de transformation publique imposait une harmonisation des temps de travail aux collectivités, avec les fameuses « 1 607 heures ». Aujourd’hui, nous savons, grâce au PLF 2024, que 83 % des communes ont appliqué cette réforme.

Ce n’est pas très différent en matière de rémunérations. Bien sûr, les récentes hausses du point d’indice sont tout à fait nécessaires face à l’inflation, plus encore que cette prime de pouvoir d’achat exceptionnelle rendue possible pour tous les agents, dont les agents territoriaux. À cet égard, comment ne pas regretter qu’il y ait eu un aussi long délai entre les annonces et la publication du décret d’application, intervenue seulement le 31 octobre 2023 ? Dans ces conditions, il est difficile, pour les collectivités, de répondre rapidement aux revendications légitimes de leurs agents territoriaux, mais aussi de prévoir sereinement les impacts sur les budgets locaux 2023 ou 2024. Quant à la protection sociale dans la fonction publique, elle n’est pas non plus sans poser quelques problèmes. Alors que le Gouvernement affichait la réforme des retraites comme une garantie pour l’avenir des pensions, les données du PLF 2024 soulignent que, pour la troisième année consécutive, la régime de retraite des fonctionnaires devrait être déficitaire et que cela ne devrait pas s’améliorer, puisque le solde est estimé à –4,6 % en 2026. Faute d’encourager suffisamment l’emploi des fonctionnaires pour équilibrer entrées et sorties, il reviendra encore à l’État d’assurer le paiement des pensions de ses anciens agents, en augmentant significativement sa contribution employeur, donc le budget afférent.

de deux jours de carence supplémentaires pour les fonctionnaires. Le progrès social et la santé publique doivent conduire, pour les travailleurs des secteurs publics et privés, à un alignement par le haut plutôt que par le bas. J’en viens enfin aux conditions de travail de nos agents au parc immobilier de l’État et aux cités administratives, question abordée dans la mission « Transformation et fonction publiques ». Comme le rapporteur spécial a pu le souligner, on note un délai important entre les annonces et la rénovation énergétique des bâtiments concernés. Au delà des enjeux de pilotage opérationnel auxquels ils renvoient, ces délais reflètent les difficultés intrinsèques des rénovations lourdes qui touchent le patrimoine immobilier de l’État, comme celui des collectivités et des particuliers. J’attire l’attention du Gouvernement sur les leçons à tirer de ces difficultés dans la manière dont il accompagne et finance les rénovations. face à l’urgence climatique ? Peut être les démarches opérationnelles devraient elles être simplifiées ? Pour conclure sur la fonction publique et la manière de la rendre à nouveau intéressante et valorisante aux yeux de nos concitoyens, je veux dire un mot sur la formation,

limiter le nombre de contrats aidés, en raison du désengagement soudain de France Compétences, qui vient s’ajouter à l’incertitude qui pesait déjà sur la pérennité du soutien de l’État. Cette situation est d’autant plus injuste qu’elle crée un décalage entre employeurs privés et publics. Aussi proposerons nous un amendement de 5 millions d’euros à destination du CNFPT visant à compenser la baisse de participation de France Compétences. Nous soutiendrons les autres initiatives permettant de pérenniser la participation de l’État en la matière.

Il sera malheureusement difficile d’aller beaucoup plus loin, car la présence territoriale des services des impôts ou des douanes est indispensable pour les citoyens, les acteurs économiques et les collectivités locales.

Dans quelle mesure un suivi des absences ne serait il pas jugé discriminatoire ou attentatoire au secret médical ? L’alignement du jour de carence est une étape. Pour le rendre pleinement effectif, il faudra aussi, à terme, distinguer les fonctions d’assureur et d’employeur dans la fonction publique. Concernant les effectifs, le rapporteur spécial soulève avec justesse la question de la réserve opérationnelle des douanes. Cette dernière n’est pas prête, alors qu’elle devait apporter un renfort utile dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Au delà des douanes, la question de la gestion des ressources humaines va se poser dans plusieurs pans de la fonction publique, à l’occasion de cet événement

D’ailleurs, près de 590 millions d’euros de crédits sont ouverts à ce titre pour 2024. Malheureusement, Bercy n’échappe pas à la malédiction des projets informatiques publics. Les coûts de tous les projets sont révisés à la hausse et les dates de livraison sont décalées.

Le ministère de l’économie, qui abrite la direction de l’immobilier de l’État, devrait être le fer de lance des politiques ministérielles. C’est vrai ! Je relève avec malice que le retard pris pour la rénovation des cités administratives a permis de tenir compte des évolutions des modes de travail à la suite de la crise de la covid 19 et du recours accru au télétravail, avec un impact notable sur la gestion des surfaces des bâtiments. Cela ne vous a d’ailleurs pas échappé, monsieur le ministre. Vos annonces du 21 novembre dernier

Je comprends que l’État ait envie de se débarrasser de quelques passoires thermiques : il n’y a pas de temps à perdre pour respecter le calendrier exigé par le décret tertiaire de la loi portant Il s’agit là d’un chantier énorme, pour lequel l’État a déjà dépensé 3,9 milliards d’euros sur les trois dernières années. C’est un chantier « pharaonique », considéré comme « le chantier du siècle » par le ministre de la transition écologique, Christophe Béchu.

les prix de l’immobilier baissent depuis plusieurs mois : la période actuelle n’est donc peut être pas la meilleure pour vendre les bijoux de famille. Enfin, l’idée de créer une foncière et d’instaurer des loyers pour chaque ministère n’est pas nouvelle

2020. Avant de conclure, je ne peux manquer de partager l’inquiétude de la rapporteure spéciale Sylvie Vermeillet quant à la croissance inéluctable du déficit du régime de retraite des fonctionnaires d’État. En effet, celui ci atteindra 2,5 milliards d’euros Du fait du gel du point d’indice pendant de nombreuses années et de la revalorisation limitée de ces deux dernières années, les salaires des fonctionnaires augmentent moins vite que les pensions, qui vont connaître une hausse de 5,2 %, pour la retraite de base, en janvier 2024.

Une note très intéressante de Jean Pascal Beaufret, présentée lors de la réunion du Conseil d’orientation des retraites qui s’est tenue le 21 septembre dernier, dénonce l’absence d’identification du solde des caisses de retraite dans l’ensemble des administrations de sécurité sociale.

compte tenu de l’absence de caisses de retraite juridiquement séparées, transforme profondément les comptes nationaux. La majoration de 33 % des rémunérations des personnels de l’État par une importante subvention d’équilibre augmente le PIB en conséquence. Dans le même temps, les prélèvements obligatoires sont réduits par rapport à des cotisations effectives. Pour conclure, je ne saurais dire mieux que M. Beaufret : « Pour les comptes de la Nation comme pour les comptes de l’État, des méthodes légales, fondées sur le choix de taux de cotisation exorbitants du droit commun et non pas sur celui “d’un pourcentage raisonnable des salaires versés aux personnels en activité”, ne vont donc pas dans le sens d’une transparence des comptes publics.

la réforme des retraites a marqué le débat public en 2023. Elle déploie désormais ses premiers effets. C’était une réforme courageuse, que le Sénat a votée en responsabilité. Ce qui n’est pas responsable, c’est de laisser croire aux Français que la retraite à 60 ans ou 62 ans serait un acquis social ou un droit inaliénable, alors que les évolutions démographiques ébranlent l’équilibre de notre régime de retraite – nous l’avons entendu et compris. Le relèvement à 64 ans de l’âge légal de départ à la retraite est un effort important pour nombre de nos concitoyens. Mais les scénarios du COR sont clairs : ces efforts ne seront pas suffisants pour assurer le financement du régime à long terme. Ainsi, dès 2027, le système de retraite présentera un déficit à hauteur de 0,3 % du PIB, déficit qui ne cessera de se creuser au cours des prochaines décennies. Or ces chiffres n’intègrent pas le régime de retraite des fonctionnaires. En effet, les dépenses liées au versement des pensions sont comptabilisées non pas dans le budget de la sécurité sociale, mais dans le budget général, et précisément dans la mission « Régimes sociaux et de retraite », que nous examinons aujourd’hui. est pourtant colossal : en y ajoutant le compte d’affectation spéciale « Pensions », le montant global de ces crédits atteint 74 milliards d’euros. C’est plus d’un quart des pensions de retraite versées par les régimes de base. Ces pensions sont financées non par les cotisations des assurés, mais par l’impôt. On pourrait dire que c’est du pareil au même, puisque les impôts, comme les cotisations, sont des prélèvements obligatoires. Mais cette différence pose un problème de fond, qui tient à la lisibilité de notre système de retraite. Il faut dire les choses clairement : l’équilibre de notre régime dépend de la solidarité nationale. Cela vaut tout particulièrement pour les régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP. Tous deux ont été fermés, mais, en vertu de la clause dite du « grand père », ils continuent d’être financés par la solidarité nationale pour tous les salariés qui étaient employés avant la réforme. Ces deux régimes représentent plus de 70 % des subventions d’équilibre des régimes spéciaux. Au total, cette dépense représente plus de 6,2 milliards d’euros. Il nous semble plus pertinent de conserver le schéma de financement actuel, afin de garder un suivi précis du coût de ces régimes pour nos finances publiques. Avant de terminer, je souhaite évoquer la mission « Gestion des finances publiques », qui regroupe les crédits alloués à Bercy. En 2024, le schéma d’emplois serait stabilisé, après plusieurs années de réduction des effectifs. Notre groupe tient à saluer les efforts qui ont été réalisés pour rationaliser ces effectifs. Bercy a prouvé que l’on pouvait faire mieux avec moins. Ses services sont largement reconnus comme particulièrement performants et efficaces au sein de notre administration. Pourtant, cette qualité de service n’implique pas une hausse continue des effectifs. C’est peut être un exemple à suivre. collègues, notre groupe avait proposé une réduction globale du schéma d’emplois des effectifs de l’État, à hauteur de 5 % sur l’ensemble du quinquennat. Le Sénat avait adopté cette proposition. Le Gouvernement n’a intégré cet objectif ni dans la loi de programmation ni dans le projet de loi de finances. Il s’agit pourtant d’une étape indispensable pour engager le désendettement de l’État.

aussi le terrorisme et le trafic d’êtres humains. Elle séduit, parce que ces activités criminelles rapportent beaucoup d’argent aux organisations terroristes : là où le trafic de produits stupéfiants rapporte 200

Les sujets traités ne sont pas des moindres : immobilier de l’État, administration fiscale, pensions de retraite. Pour tout cela, nous avons droit à quarante cinq minutes de discussion générale et deux heures quinze Dans ce contexte, il ne faut pas s’étonner du décalage entre l’importance de nos travaux en séance publique et l’intérêt de nos concitoyens. Ce que nous nous apprêtons à faire cet après midi y contribue grandement ! Sur le fond, trois grands sujets se détachent de cette séquence. Tout d’abord, l’immobilier de l’État. Ne nous y trompons pas, le compte d’affectation spéciale du même nom ne représente qu’une petite partie de l’ensemble du patrimoine immobilier de l’État : il fait état d’un montant de 340 millions d’euros sur une valeur comptable estimée à 73,3 milliards d’euros, donc seulement 13 % des dépenses d’investissement de l’État en la matière. Ce compte, destiné à abonder les entités et ministères qui auraient mutualisé leurs produits de cession, n’est manifestement qu’un gadget comptable à l’intérêt plus que limité. La question de son maintien se pose dès lors clairement et j’aimerais que l’on m’explique ce qu’il apporte en lisibilité et en efficacité à une discussion budgétaire déjà bien complexe. Ce n’est

a là un véritable enjeu. Les montants encaissés au titre du contrôle fiscal s’élèvent à 10,6 milliards d’euros pour 2022, un chiffre rigoureusement identique à celui de 2021. Ce n’est pas satisfaisant

de récupérer ces sommes importantes dont nous avons bien besoin. Ce n’est visiblement pas la direction que compte prendre la majorité sénatoriale. En effet, au sein de la mission « Transformation et fonction publiques », qui traite aussi de tous les emplois de l’État et de ses opérateurs, le rapporteur général va proposer une baisse indifférenciée

Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, ce projet de loi de finances pour 2024 devait concrétiser les annonces de l’ancien ministre du budget, M. Gabriel Attal, en matière de lutte contre la fraude fiscale.

Ce budget prévoit d’ailleurs de renforcer les moyens technologiques au détriment des moyens humains. Les contrôles sur place s’effondrent depuis 2013, et c’est la lutte contre la fraude fiscale qui en pâtit, car elle représente 30 % de cette modalité de contrôle.

le Conseil des prélèvements obligatoires (CPO) expliquait que cette stratégie de baisse des moyens « aurait dû se traduire par un meilleur ciblage des contrôles et une réduction du nombre d’affaires à faible rendement et d’affaires conformes ».

Nous attendions avec impatience ce débat pour dévoiler la supercherie qui consistait à annoncer, lors de la présentation du plan Fraude, un renforcement sans précédent des moyens,

donc un amendement visant à engager un vaste plan de recrutement de contrôleurs fiscaux : 500 cette année, 500 l’année prochaine et 500 l’année suivante. Pas de tour de passe passe ! Les personnels méritent mieux que des annonces tronquées

Nous sommes, par exemple, le deuxième domaine maritime mondial après les États Unis. Le contrôle et la surveillance d’espaces maritimes de plus de 10 millions de kilomètres carrés mériteraient au moins une flotte sérieuse, afin de permettre aux quelques agents des douanes disséminés aux quatre coins du monde d’assumer réellement

au travers de quatre missions substantielles et de deux comptes spéciaux non moins déterminants. C’est bien peu ! Vous me pardonnerez donc d’avance de ne pas être exhaustif. Au nom du groupe RDSE, je m’autoriserai à effectuer des choix et, comme nous le disons à Marseille, à aller droit au but. Tout d’abord, je veux évoquer la mission « Gestion des finances publiques », dotée d’une enveloppe proche de 11 milliards d’euros. Très sommairement, je m’attellerai à rappeler les moyens alloués pour poursuivre et finaliser la modernisation de la

Je pense notamment à la technique de la fouille de données que l’on nomme plus communément – utilisant un affreux anglicisme –, et au programme de mobilité Télémac pour cibler avec efficience les contrôles, dont le produit est évalué à près de 10 milliards d’euros. J’ai aussi à l’esprit le portail Chorus factures, qui s’adresse aux entreprises pour une meilleure facturation interentreprises. Ensuite, comment ne pas parler ici des collectivités territoriales, en se félicitant de la poursuite de l’expérimentation du compte du compte financier unique ? Celui ci a pour objectif de rendre lisible la production des états comptables et devrait être pérenne d’ici à 2027. Je veux aussi évoquer la mission « Transformation et fonction publiques », qui connaît, quant à elle, une hausse de 379,5 millions d’euros par rapport à 2023 pour atteindre 1,2 milliard d’euros. On se félicitera des actions tendant à rendre la fonction publique attractive ; à lutter contre la crise du du sens apparue chez nos serviteurs de l’État ; à juguler la déperdition des talents vers le secteur privé. Ces trois objectifs appellent une mobilisation constante afin de redonner du muscle et du tonus à notre service public. L’effort devrait être plus marqué, mais, disons franchement, il donne tout de même une orientation ! Dans cette perspective, je me réjouis de la mise en orbite de la complémentaire santé à l’horizon de 2026 et des contrats de prévoyance à compter du 1 janvier 2025 – réformes tant attendues par les agents.

La fidélisation des agents passe aussi, au travers du programme 348, par une offre d’un environnement professionnel de qualité, grâce au lancement d’une nouvelle séquence de rénovation énergétique des bâtiments de l’État. Enfin, il m’importe de ne pas passer sous silence les crédits non répartis, c’est à dire les crédits dont la dépense est difficilement prévisible. Une question, messieurs Quelle suite réserverez vous à la demande de bilan formulée par la Cour des comptes, en mai dernier, sur le recours systématique au programme 551 pour financer des décisions prises lors des rendez vous salariaux annuels

pour examiner conjointement les missions « Transformation et fonction publiques », « Gestion des finances publiques », « Crédits non répartis » et « Régimes sociaux et de retraite ». Dans un souci de concision, je vais souligner brièvement les points clés de chaque mission. Les missions « Gestion des finances publiques » et « Transformation et fonction publiques poursuivent la dynamique engagée depuis 2017 pour moderniser notre action publique et transformer notre administration, tout en améliorant la qualité des services publics. La mission « Gestion des finances publiques », qui inclut la DGFiP et la direction générale des douanes et droits indirects maintient en 2024 un niveau élevé de crédits, après l’augmentation notable de 2023 qui avait marqué une rupture avec la tendance antérieure. Le groupe RDPI se réjouit de l’amplification des actions de lutte contre la fraude et de contrôle, avec le recrutement prévu de 1 500 agents supplémentaires d’ici à 2027 pour renforcer les équipes de la DGFiP.

Nous saluons également la modernisation des espaces de travail dans le cadre de la stratégie immobilière en cours, démontrant un engagement fort envers la transition écologique et la réduction de l’empreinte carbone. La mission « Transformation et fonction publiques », notamment le programme 349, contribue à inverser la dynamique à inverser la dynamique de rupture des Français avec leur administration, pour des services plus accessibles et plus proches. Le groupe RDPI soutient les efforts visant à renforcer l’attractivité de la fonction publique, notamment avec la poursuite du programme « Fonction Publique + ». Concernant la mission « Régimes sociaux et de retraite », soulignons le contexte particulier marqué par l’entrée en vigueur en septembre 2023 de la réforme paramétrique des retraites. Malgré des économies réalisées, la réforme n’aura pas d’effet avant 2025 sur les principaux régimes spéciaux bénéficiaires des crédits de cette mission, à savoir ceux de la SNCF et de la RATP. Avec 6,2 milliards d’euros, cette mission demeure cruciale pour le versement des pensions de milliers d’affiliés. En ce qui concerne la mission « Crédits non répartis », la hausse significative des crédits du programme 551, consacrée principalement aux évolutions statutaires de la couverture de prévoyance des agents publics de l’État, contraste avec la baisse conséquente du programme 552, rompant avec les années de crise sanitaire. En conclusion, ces missions du PLF 2024 représentent des avancées substantielles dans la modernisation de notre administration, la gestion financière de l’État et la soutenabilité de nos

pourquoi je vous propose de profiter de cet examen budgétaire pour présenter mes priorités d’action au travers des quatre programmes structurants composant le budget du ministère.

pourvoyons de 250 emplois supplémentaires dès cette année, tout en continuant à redéployer des postes et à tirer parti de la numérisation, ce qui permet une réduction nette de 200 effectifs. Ce budget est donc cohérent avec notre double objectif de modernisation de l’administration fiscale et de lutte contre toutes les fraudes, le tout en maintenant un haut niveau de service qui fait, je crois, de la DGFiP et de ses implantations l’un des services publics préférés des Français. Nous renforçons également les effectifs dédiés aux renseignements douaniers et ceux de Tracfin pour la détection des flux financiers illicites. La douane déploiera de nouveaux effectifs pour mieux surveiller nos frontières ; ses moyens d’investigation et ses équipements seront modernisés. Pour ce qui concerne les autres points d’attention soulevés par le rapporteur je me félicite du déploiement du nouveau réseau de proximité de la DGFiP, ainsi que de la qualité du travail des conseillers aux décideurs locaux auprès des collectivités territoriales. Sur le sujet de la transition écologique, j’entends le scepticisme qui s’exprime au regard de la multiplication des démarches vertes

la consommation d’énergie des bâtiments a diminué de 13 % en 2022 ; une sortie totale des chaudières au fioul est prévue d’ici à 2025. Ces évolutions s’expliquent par des investissements importants et nécessaires du ministère.

Le montant de la première s’explique notamment par l’incertitude sur la ventilation des volets santé et prévoyance de la réforme de la protection sociale complémentaire des agents publics de l’État. La seconde connaît une diminution sensible de crédits par rapport à 2023. La commission des finances souhaite réduire davantage le montant de ces deux dotations. Nous pensons toutefois que l’État a le devoir d’être prévoyant, sachant que ces crédits pourront naturellement être annulés en cours d’exercice compte tenu des informations disponibles.

Je veux également dire un mot du programme 348, consacré à la performance et à la résilience des bâtiments de l’État. Conformément aux engagements pris dans le cadre de la planification écologique, 550 millions d’euros supplémentaires seront engagés en 2024 sur la base d’un appel à projets

Comme j’ai eu l’occasion de l’indiquer lors de l’examen du PLFSS, la trajectoire de solde, bien que toujours déficitaire, s’améliore sous l’effet de la réforme des retraites, en particulier la réduction du flux de nouveaux retraités. Ainsi, à l’horizon de 2027, le déficit sera inférieur de 6 milliards d’euros à ce qu’il aurait été en l’absence de réforme. Ce n’est pas une

en diminuant l’enveloppe ouverte sur le programme 349 « Transformation publique ». En effet, si la programmation des crédits de ce programme a toujours été ambitieuse au cours des dernières années, l’exécution s’est rarement montrée à la hauteur des objectifs affichés, avec d’importants retards constatés sur le décaissement des crédits. Au 30 octobre 2023, les montants de crédits de paiement consommés sur le programme 349 s’élevaient ainsi à 122 millions d’euros, contre 251 millions pour 2023. Pourtant, le présent projet de loi de finances prévoit pour 2024 de nouveaux montants très élevés pour ce programme, et plus particulièrement 140 millions d’euros pour l’action n° 01 « Fonds pour la transformation de l’action publique ». Une mesure de sincérisation apparaît donc nécessaire.

L’avis de la commission est doublement défavorable

de la mission « Économie », dont les crédits ont déjà été adoptés par le Sénat. Très bon argumentaire ! Ensuite, sur le fond, le partage du financement de la rémunération des conseillers, tel qu’il est prévu dans le cadre du conventionnement de la subvention versée par l’État aux structures employant ces derniers, apparaît équilibré.

comprend bien une dotation budgétaire de 15 millions d’euros au titre de l’apprentissage dans la fonction publique territoriale. L’annexe budgétaire précise que ces crédits seront versés sous forme de subvention au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) : votre objectif est donc atteint. L’amendement étant satisfait,

pour la fonction publique et l’inscrire dans nos politiques de recrutement et de ressources humaines. L’engagement avait été pris de consacrer 15 millions d’euros aux lignes budgétaires de mon ministère pour accompagner et financer l’apprentissage dans les collectivités territoriales.

le maintien de ces 15 millions d’euros sur les trois années à venir, pour éviter tout effet de retrait de l’État dans la politique d’apprentissage à destination des collectivités territoriales. Nous avons traduit cet engagement en signant récemment

Cet indicateur ne permet pas de connaître le coût de gestion des prestations d’action sociale, dont la maîtrise demeure tout de même un enjeu important, et ne porte que sur le chèque emploi service universel pour la garde des enfants de moins de 6 ans. Il est difficile d’en tirer des enseignements, dans la mesure où il atteint depuis sa création un taux très élevé de satisfaction : les marges de progression sont très faibles. Cet amendement vise donc à remplacer cet indicateur par les deux indicateurs qui étaient posés auparavant le coût de gestion des prestataires extérieurs chargés de la gestion de certaines prestations d’action sociale et le coût moyen annuel de réservation d’une place en crèche. L’amendement

la consultation d’une fiche n’est pas en tant que telle signe de l’attractivité d’un poste. D’autre part, la cible, fixée à vingt candidats pour les trois prochaines années, semble peu ambitieuse. Je vous propose de le remplacer par un indicateur visant à mesurer le taux du nombre de candidatures reçues pour une fiche de poste publiée par rapport au nombre de consultations de cette même fiche. Ainsi, il sera possible de savoir dans quelle mesure la consultation d’une fiche se traduit effectivement par le dépôt d’une candidature, ce qui contribuera à évaluer l’attractivité du poste et, plus

La droite tient au respect des traditions. Et s’il en est une qu’elle n’abandonnerait pour rien au monde, c’est bien celle qui la conduit à accuser la fonction publique d’être budgétivore.

un peu plus d’un employé sur cinq – 21 % précisément – travaille dans la fonction publique. Si ce chiffre est supérieur à la moyenne des pays européens de l’OCDE, qui se situe à 19 %, pays est loin d’être celui qui compte le plus d’agents publics en proportion de l’emploi total. En Norvège, près d’un salarié sur trois, soit 31 %, est employé dans le secteur public. Le ratio est de plus d’un salarié sur quatre en Suède, soit 29 %, et au Danemark de 28 %. Plutôt que de réduire aveuglément le nombre de fonctionnaires, le débat devrait se concentrer sur l’amélioration de l’action publique, les modes de recrutement, la rémunération et la gestion des carrières du secteur public. Se focaliser ainsi sur les chiffres sans mettre en face les missions d’intérêt général que l’on assigne aux fonctionnaires appauvrit le débat. Surtout, je note que vous ne précisez pas quels secteurs seront affectés par ces suppressions de postes.

se justifierait par l’existence de nombreux doublons dans les missions assumées par les opérateurs de l’État et d’autres entités, en particulier les collectivités territoriales… Je rappelle que les opérateurs qui mobilisent les subventions pour charges de service public les plus importantes dans le PLF pour l’an prochain sont : les universités pour 12,3 milliards

L’article 115 de la loi de finances pour 2018 a réinstauré un jour de carence dans la fonction publique. L’évaluation préalable de cet article estimait alors l’économie supplémentaire liée à la réinstauration d’un jour de carence à 108 millions d’euros, et à 216 millions d’euros en cas d’extension du délai de carence à trois jours. Compte tenu du dynamisme des effectifs de la fonction publique d’État depuis 2018, cette économie est désormais estimée à 220 millions d’euros pour l’année 2024. Par convention, cette économie est imputée sur le programme 551, « Provision relative aux rémunérations publiques », de la mission « Crédits non répartis », à hauteur de 220 millions d’euros en autorisations d’engagement et en crédits de paiement. il ne s’agit pas de remettre en cause les mesures financées par la provision relative aux rémunérations publiques en 2024. L’économie réalisée grâce aux dispositions de cet amendement a en effet vocation à être répartie dans l’ensemble des missions du budget de l’État. Je rappelle que cet amendement a déjà été adopté par le Sénat

en ce qui concerne l’année 2023, seuls 20 millions d’euros de crédits ont été consommés à ce jour, soit 2 % des crédits ouverts. Par ailleurs, les montants demandés en 2024 demeurent sensiblement supérieurs aux montants conventionnels de 424 millions d’euros

le ministre délégué. Les fonctionnaires de La Poste et d’Orange peuvent accéder à des dispositifs de préretraite. En l’état actuel du droit, ils peuvent cumuler le dispositif de préretraite de leur employeur et le dispositif de retraite progressive de la fonction publique.

qui ont pour objectif d’aménager la réduction ou la cessation d’activité des salariés en fin de carrière. Orange, en particulier, a mis en place un système de préretraite d’entreprise appelé « temps partiel senior », qui permet à ses employés de réduire leur temps de travail tout en conservant une partie de leur rémunération. Selon les estimations

préretraite d’entreprise prévu par l’article 96 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024. Par conséquent, la commission émet un avis favorable sur cet amendement, qui précise utilement que le dispositif de retraite progressive des fonctionnaires est exclusif d’une préretraite d’entreprise.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le montant global des crédits demandés dans le cadre du présent projet de loi de finances pour la mission « Culture s’élève cette année à plus de 3,8 milliards d’euros en crédits de paiement, mais atteint 4,1 milliards d’euros en autorisations d’engagement, soit une forte progression par rapport à l’année dernière.

très significative. Ainsi, 230 millions d’euros avaient été accordés dans le cadre du plan de relance au secteur du spectacle vivant. La fin de ces crédits exceptionnels ne signifie pas pour autant celle des inquiétudes pour l’ensemble de ce secteur, confronté à un effet budgétaire de ciseaux entre la reprise de l’activité et la progression du coût des dépenses contraintes, notamment en matière d’énergie. Une part non négligeable des nouveaux moyens accordés en 2024 vise à compenser une partie de la hausse de ces dépenses. Ainsi, 41 millions d’euros sont prévus pour les opérateurs du patrimoine, particulièrement affectés par le renchérissement des matériaux de construction, qui touche

une réduction des marges artistiques, les établissements étant amenés à revoir leur programmation afin de diminuer les coûts de production des spectacles. Une interrogation demeure incidences des jeux Olympiques et Paralympiques, qui devraient contraindre certains lieux à fermer et certains festivals à être décalés. Au delà de ces questions, les crédits du programme 131 sont stabilisés après la hausse enregistrée l’année dernière. Je note cependant l’abandon

Pierrefitte sur Seine. Concernant Beaubourg, les travaux nécessaires priveront le musée de ressources propres pendant les quatre ans de fermeture complète. Si le montant du projet est actuellement estimé à 262 millions d’euros, il est à craindre que l’inflation n’entraîne une augmentation de la facture.

Sa réalisation a été permise grâce aux crédits du plan de relance. Au vu des efforts consentis dans ce budget, notamment en faveur du patrimoine, et tout en gardant à l’esprit certains points d’alerte, la commission des finances propose d’adopter les crédits de la mission.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, en complément des propos de mon collègue rapporteur spécial, je me concentrerai sur les programmes 224 et 361, qui comprennent les crédits liés à l’éducation artistique et culturelle, à l’enseignement supérieur culturel et aux moyens de fonctionnement du ministère de la culture. Ce projet de loi de finances prévoit de majorer la dotation du programme 361 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », de près de 4 % en autorisations d’engagement et de 3,6 % en crédits de paiement par rapport à 2023 ; ces crédits devraient ainsi atteindre environ 830 millions Sur ce montant, les sommes allouées aux établissements d’enseignement supérieur culturel et à l’insertion professionnelle devraient progresser de 23 millions d’euros en crédits de paiement, afin de répondre à différents objectifs. Tout

nous pouvons nous féliciter. La contribution du ministère en faveur de ces écoles devrait atteindre 218 millions d’euros en crédits de paiement. Leur plafond d’emplois devrait en outre être relevé de trente équivalents temps plein.

prévus pour le financement du pass Culture. Je constate donc une certaine stabilité des moyens par rapport à l’année précédente. Il faut toutefois noter que les crédits accordés par le ministère de l’éducation nationale pour le financement du volet collectif du pass Culture sont quant à eux en hausse. est aujourd’hui le deuxième opérateur du ministère de la culture, juste derrière la Bibliothèque nationale de France. Avec mon collègue Vincent Éblé, nous avons consacré au pass Culture un travail de contrôle budgétaire

Au delà du pass Culture, les crédits affectés à l’éducation artistique et culturelle sont stables et s’élèvent à 180 millions d’euros. Contrairement aux craintes parfois formulées, le déploiement du pass Culture ne semble pas avoir entraîné de diminution des moyens de l’éducation artistique et culturelle Cet outil a donc vocation non à se substituer aux dispositifs existants, mais plutôt à les renforcer, en ciblant des publics parfois différents. J’en viens maintenant au programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture », qui devrait être doté de plus de 810 millions d’euros en 2024. Ce programme regroupe l’ensemble des dépenses de personnel des agents directement rémunérés par le ministère de la culture. lors de l’exercice précédent, la masse salariale devrait croître en 2024 et atteindre 539 millions d’euros. Cela représente une hausse de 4,9 %, soit 26 millions d’euros, par rapport à 2023. Une partie importante de cette augmentation découle de mesures générales : les hausses successives du point d’indice en 2022 et en 2023, l’octroi de cinq points d’indice supplémentaires à l’ensemble des agents au 1 janvier 2024, la revalorisation des jours de congé du compte épargne temps et, enfin, la prise en charge à 75 des frais de transport. L’ensemble de ces mesures représente un montant global de 6,2 millions d’euros. Ces évolutions sont bienvenues ; elles démontrent la prise en compte des difficultés des agents dans le contexte de forte inflation que nous connaissons. À cela s’ajoutent des mesures catégorielles nouvelles, pour un montant de 5,5 millions d’euros, destinées à revaloriser la rémunération des agents contractuels ainsi que le régime des enseignants chercheurs des écoles nationales d’architecture. Encore une fois, il s’agit d’une réponse forte aux difficultés de ces écoles, difficultés qui avaient été soulignées au cours de plusieurs mouvements sociaux en début d’année. Enfin, le programme 224 devrait également supporter une partie des coûts exceptionnels liés au financement de l’opération Capitale européenne de la culture de 2028, pour laquelle quatre villes ont été présélectionnées par le jury européen : Montpellier, Bourges, Clermont Ferrand et Rouen.

C’est pourquoi la commission de la culture se réjouit que les crédits de l’État en faveur des patrimoines progressent une nouvelle fois l’année prochaine ; même si cet effort financier ne compensera pas la hausse des coûts, il permettra d’en atténuer les effets et d’inscrire la protection du patrimoine dans la durée. sans nier la nécessité des grands projets du centre Pompidou et des Archives nationales à Pierrefitte sur Seine, la commission de la culture s’inquiète de la faiblesse des marges de manœuvre qui subsisteront pour les chantiers à mener au cours des années à venir dans les territoires, chantiers essentiels à leur développement et à leur attractivité. Il est vrai que l’État contribue aussi de plus en plus, par des leviers fiscaux, à stimuler la générosité publique en faveur de la cause du patrimoine. La commission de la culture se félicite des mesures prises en faveur du patrimoine religieux des petites communes après les alertes lancées voilà un an et demi par nos par nos collègues Anne Ventalon et Pierre Ouzoulias. Nous serons très attentifs à leur mise en œuvre et nous espérons que le volet « ingénierie » de ces mesures pourra être complété, tant il s’agit d’un enjeu crucial pour les collectivités, très démunies dans ce domaine. La commission est en effet convaincue que c’est en accompagnant mieux les collectivités sur le plan technique que nous pourrons franchir un nouveau cap en matière de préservation du patrimoine. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous plaidons avec ardeur pour le renforcement des effectifs des services déconcentrés de l’État chargés du patrimoine. le besoin d’ingénierie des collectivités ne se limite pas à la problématique du patrimoine religieux. Prenons deux exemples. Le premier a trait à l’entretien du patrimoine. Comment expliquer que les crédits destinés à l’entretien des monuments qui n’appartiennent pas à l’État soient sous consommés, alors qu’un entretien plus régulier de nos monuments profiterait à nos finances publiques à moyen terme ? Est ce lié à un problème de moyens humains ou à un déficit de pédagogie ? relatif à la rénovation énergétique du bâti ancien : malgré quelques progrès visant à mieux conjuguer l’urgence de la rénovation thermique avec la préservation du patrimoine, beaucoup reste encore à accomplir

La revalorisation des subventions des opérateurs, en particulier des services d’archéologie des collectivités territoriales, n’est pas à la hauteur de l’explosion des coûts de réalisation des diagnostics, alors même que la redevance d’archéologie préventive rapporte bien plus à l’État que ce que celui ci reverse aux services des collectivités et à l’Institut national de recherches

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, la commission de la culture se réjouit que l’État maintienne en 2024 son effort en faveur de la création ainsi que de la transmission des savoirs et de la démocratisation de la culture. Malgré la reprise de leur fréquentation, les établissements culturels restent dans une situation très fragile. La commission estime qu’il est urgent de restaurer leurs marges artistiques, faute de quoi la diversité culturelle, l’animation des territoires et l’accès à la culture de nos concitoyens pourraient être rapidement menacés. nous espérons que le plan Mieux produire, mieux diffuser permettra de répondre effectivement à l’enjeu et portera rapidement ses fruits. En ce qui concerne le budget de la création, trois sujets nous préoccupent. la situation des scènes de musiques actuelles, à propos de laquelle nous vous présenterons un amendement. Ensuite, les festivals se trouvent dans une situation délicate, compte tenu des incertitudes causées par l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Enfin,

En ce qui concerne la transmission des savoirs, la commission salue les efforts consentis pour les écoles nationales supérieures d’architecture ; cela traduit un réel progrès, même si celui ci doit être complété. Nous sommes en revanche

dans les territoires. S’il est vrai que ces écoles relèvent d’abord des collectivités territoriales, l’État doit se trouver aux côtés de celles ci pour les aider à traverser cette crise. Chaque fermeture d’école entraîne une diminution des débouchés pour nos jeunes dans l’enseignement supérieur et le maillage territorial et l’égalité d’accès à l’enseignement supérieur s’effritent. Soyons cohérents avec la priorité accordée à la jeunesse en matière de démocratisation culturelle. Le pass Culture n’atteindra ses objectifs que s’il peut s’appuyer sur l’existence d’une offre culturelle solide et diversifiée dans l’ensemble des territoires. Rappelons nous est un outil et non une politique. Pour qu’il soit pleinement opérationnel, il faut le compléter par de la médiation culturelle, travailler de concert avec les collectivités au développement et à la valorisation des offres culturelles de proximité, et améliorer l’articulation de son volet collectif avec l’ensemble de la politique d’éducation artistique et culturelle,

Comparée à l’effort pour l’accès à la culture des jeunes, la politique de démocratisation culturelle dans les territoires nous paraît manquer de vision stratégique. Il faut conclure. À terme, nous demanderons une évaluation du fonds d’innovation territoriale.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons que nous réjouir de la hausse des crédits de la mission « Culture ». Certains dispositifs sont prometteurs ; espérons que ce ne soient pas des trompe l’œil. comme je l’ai déjà souligné voilà un an, le risque est que cette hausse soit neutralisée par l’inflation, alors que nous assistons au déploiement de dispositifs ambitieux. En premier lieu, il y a bien sûr la question du patrimoine. En la matière, le soutien de l’État est indispensable.

locales. Le patrimoine de proximité à protéger est détenu à 94 % par les collectivités ou par des propriétaires privés, qui doivent être soutenus. Aidons les en mobilisant des crédits pour leurs projets. Il y a de nombreuses demandes sur le terrain, mais les soutiens sont encore limités et l’on a des difficultés à articuler les dispositifs Réfléchissons à une synergie entre toutes les aides, c’est indispensable. La politique patrimoniale doit être plus ambitieuse et toucher tous nos territoires. Madame la ministre, il existe, hélas ! un déséquilibre territorial imparfaitement corrigé et il y a trop de disparités criantes.

Je me réjouis que les fonds prélevés dans le cadre d’une collecte réalisée sous l’égide de la Fondation du patrimoine soient affectés à l’aide à l’ingénierie à destination des petites communes ayant la maîtrise d’ouvrages de biens à restaurer. Ces exemples sont à multiplier. Le loto du patrimoine doit inspirer d’autres initiatives.

Sans oublier le nécessaire soutien public, il faut encourager, encore et encore, la diversification des financements, dans le prolongement des solutions proposées par mes collègues Anne Ventalon et Pierre Ouzoulias dans leur rapport Dans le domaine de l’expertise patrimoniale internationale, notre savoir faire jouit d’une image d’excellence, grâce à la formation développée dans nos structures – nos écoles d’art, l’Institut du patrimoine et tant d’autres que je ne peux citer

En ce qui concerne le spectacle vivant et les festivals, un point de vigilance s’impose, en particulier sur le sujet du rééquilibrage entre une politique de l’offre et une meilleure diffusion des crédits. Si le spectacle vivant est bel et bien de retour et que le public est de nouveau présent, il faut donner des garanties et une meilleure visibilité aux différents acteurs. La situation des scènes de musiques actuelles est inquiétante, la rapporteure l’a souligné. Les marges artistiques se réduisent et les charges augmentent. Nous restons évidemment ouverts à l’accompagnement différencié que vous avez proposé, mais nous serons très vigilants quant à son financement. Nous saluons cependant différentes mesures, comme la revalorisation du fonds festivals, mais aussi les mesures d’accompagnement spécifiques au contexte de l’année 2024, les inquiétudes s’accroissent à l’approche des jeux Olympiques et Paralympiques. Madame la ministre, nous avons besoin de signes forts : les organisateurs redoutent des annulations de dernière minute en raison de mobilisations destinées à assurer la sécurité des Jeux. Nous serons attentifs à l’indemnisation des festivals qui auront subi des pertes de recettes en raison des Jeux, sans engendrer, je l’espère, un excès de bureaucratie et de frustrations. Le modèle économique des festivals, déjà fragilisé par la crise sanitaire, est en jeu. Je me permets donc, madame la ministre, de relayer de nouveau les appréhensions des organisateurs. Toutefois, tout ne doit pas être à la seule charge des pouvoirs publics on aider les festivals à repenser leur organisation et leur financement ? J’aimerais connaître votre ambition sur ce sujet, car cette réflexion doit être partagée avec les acteurs de ce secteur. Il y a enfin l’accès à la culture, enjeu capital, en particulier pour les jeunes. L’accès à la culture reste toujours délicat.

Alors que des crédits importants sont mobilisés, comment faire en sorte que le pass Culture puisse réellement et efficacement entraîner des usages, sans recourir à la politique du carnet de chèques ? Comment faire en sorte qu’il soit un outil d’excellence, qui révèle des vocations et de futurs talents ?

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les aides exceptionnelles accordées aux acteurs de la culture pendant la crise sanitaire ont permis à ces derniers de surmonter tant bien que mal leurs difficultés.

Nombre de structures sont confrontées à des charges fixes en forte augmentation. Dans ces conditions, leur capacité à mener à bien leurs activités de création et de diffusion est fortement compromise. Un véritable risque pèse sur la programmation et l’emploi dans la filière culturelle, avec toutes les conséquences que cela impliquerait du point de vue de l’animation culturelle des territoires et de l’accès à la diversité artistique. Les établissements labellisés sont tout particulièrement fragilisés par la crise inflationniste. C’est le cas des scènes de musiques actuelles et du secteur des arts visuels, qui sont en train de connaître une véritable dévitalisation. Les soutenir plus fortement, comme le propose la commission de la culture au travers de plusieurs amendements sur cette mission, est une nécessité absolue. L’effort budgétaire de l’État en faveur de la création et de la diffusion artistiques en 2024 est certes louable, mais je crains que les financements proposés dans ce projet de loi de finances ne soient pas à la hauteur des enjeux. Ils ne permettront pas de compenser comme il conviendrait la hausse généralisée des coûts subie par les structures. En ce qui concerne la démocratisation de la culture, nous devons nous réjouir du succès du pass Culture, qui permet à de nombreux jeunes de la France entière d’accéder aux biens culturels de leur choix.

je regrette simplement que beaucoup de professeurs ne soient pas assez accompagnés par des formations en éducation artistique et culturelle pour mener des projets intéressants. Permettez moi également, madame la ministre, de vous alerter sur le manque d’accessibilité de certaines pratiques pour nos élèves atteints de handicap. Le programme « Patrimoines » est, quant à lui, particulièrement bien doté dans le projet de loi de finances pour 2024, avec 1,2 milliard d’euros en crédits de paiement. Cela représente une augmentation de 8 %, que je tiens à saluer. Une part non négligeable de ces crédits est destinée au financement de grands projets d’investissement, certains en dehors de Paris, comme la restauration du grand cloître de l’ancienne abbaye de Clairvaux ou de la cathédrale de Nantes, d’autres en Île de France, comme la rénovation du centre Pompidou ou l’extension du site des Archives nationales à Pierrefitte sur Seine. Nos rapporteures pour avis se sont émues du fait que la quasi totalité des crédits ouverts en autorisations d’engagement soit destinée à des projets situés dans le périmètre de la région capitale. Il s’agit pour elles d’un point de vigilance ; pour ma part, en tant que Francilienne, je m’en réjouis… S’agissant de projets de moindre ampleur, plusieurs sites essonniens remarquables ont pu être accompagnés par la mission Patrimoine confiée à Stéphane Bern, déployée par la Fondation du patrimoine et soutenue par les services du ministre de la culture le parc Boussard à Lardy en 2020, le château de Montagu à Marcoussis en 2021, la chapelle Saint Blaise des Simples à Milly la Forêt en 2022 et les kiosques du centre hospitalier de Bligny à Briis sous Forges en 2023. Je souhaite par ailleurs évoquer le patrimoine religieux de nos petites communes rurales, un sujet qui m’est cher. Dans le droit fil du rapport d’information de nos collègues Pierre Ouzoulias et Anne Ventalon, le Président de la République a décidé un plan d’action ambitieux destiné à accélérer la restauration et l’entretien de ces édifices au cœur de nos villes et de nos villages, qui constituent une part de l’âme de la France. projet de loi accompagne cet élan avec le relèvement du taux du crédit d’impôt accordé aux particuliers. C’est une excellente mesure. Enfin, nous savons que la prévention face au changement climatique passe à la fois par la réduction de notre consommation d’énergie et par l’amélioration de ce que nous appelons désormais la performance environnementale des bâtiments. La transition écologique du bâti ancien à préserver représente un défi tout particulier, dans la mesure où il s’agit de rénover ce bâti sans porter atteinte à sa valeur patrimoniale. Je soutiens pleinement notre rapporteur pour avis, qui a déposé un amendement portant sur l’extension aux travaux intérieurs réalisés à des fins de rénovation énergétique l’avantage fiscal lié au label délivré par la Fondation du Patrimoine, qui est actuellement limité aux travaux extérieurs. extérieurs. La culture est le creuset du vivre ensemble. Les défis à relever sont immenses tant les liens sociaux semblent se déliter au sein de notre société. J’appelle donc de mes vœux une mobilisation collective pour favoriser l’accès de tous les Français à la culture et à la création, dans tous les territoires. Madame la ministre, nous vous accompagnerons dans cette voie.

perturber les programmations des saisons et des festivals. Tout coûte plus cher et la variable d’ajustement réside dans la marge artistique. Or la compensation incomplète, par ce budget pourtant en hausse, des surcoûts subis colmate difficilement les brèches d’un système dont la résistance s’émousse, sapant les bases d’un réseau culturel construit depuis tant d’années pour assurer la diversité de l’offre, des acteurs et des structures, une diversité vitale, qui apporte un ailleurs et d’autres possibles à tous les publics. Ce budget est dit « de transformation et de transition », mais il nous semble que l’urgence est surtout à la sécurisation.

Mêmes maux, mêmes effets ; autre point d’alerte : les scènes de musiques actuelles, qui peinent à s’équilibrer, au détriment du soutien à l’émergence des artistes. La commission de la culture propose un amendement visant à garantir un plancher minimal revalorisé de la part de l’État ; nous comptons sur votre soutien. Enfin, comme tous les ans, nous déplorons la place réduite réservée aux arts visuels dans ce budget. Pourtant, ils sont très présents dans nos territoires, au travers des dispositifs de monstration, des expositions, des résidences et des échanges nombreux entre les artistes et tous les publics. Ce secteur a un besoin vital d’être mieux structuré, avec un observatoire réel des pratiques, mais cela a un coût. Or seulement 10 % des crédits du plan Mieux produire, mieux diffuser leur sont consacrés. Nous soutenons la proposition de la commission visant à augmenter cette aide, en écho à leur rôle majeur, à l’échelon tant local que national.

Bref, le compte n’y est pas… Pour terminer, abordons le budget du programme « Patrimoines », qui connaît une croissance substantielle. Pourtant, il creuse, en quelque sorte, les failles des budgets précédents. Nous attendons encore un ministère stratège en matière de patrimoine. Le fait d’orienter presque tout sur les opérateurs et le patrimoine classé ou inscrit de l’État n’exonère pas d’avoir une vision globale et d’accompagner le le reste. Prenons en exemple l’un des objectifs phares du ministère : les églises et les bâtiments cultuels présents dans toutes nos communes. Dans leur excellent rapport, nos collègues Anne Ventalon et Pierre Ouzoulias avaient identifié ces bâtiments comme prioritaires et nécessitant un plan global d’accompagnement. Qu’en

Je termine par les crédits d’entretien, essentiels pour éviter les atteintes graves au bâti. Les crédits dans ce domaine ne bougent pas, malgré nos alertes répétées des dernières années. Pis, il y a une forte sous consommation des crédits destinés aux monuments historiques n’appartenant pas à l’État.

Quelque 500 tonnes de ce métal ont été déposées en plein cœur de la capitale, au sommet de Notre Dame, pour reconstituer la croix de la flèche de l’édifice. de l’incendie tragique de la cathédrale, le dépôt de ce matériau toxique sur les trottoirs, dans les jardins et dans les cours d’école a bouleversé la vie des riverains. Ma collègue Anne Souyris a fait de cette chape son combat.

encore incertaine. Pourquoi ne pas l’utiliser pour envisager une solution architecturale plus respectueuse de la santé publique ? Le pape a été également

À quoi sert l’impôt s’il ne contribue pas à entretenir nos bâtiments publics ? Imagine t on couvrir de publicités les églises pour en financer la rénovation des toitures ? Je m’inquiète également de la surreprésentation des projets parisiens dans les investissements du ministère. C’est le cas de la rénovation du centre Pompidou, comme l’a souligné notre collègue rapporteur Sabine Drexler, dont je salue le travail.

Après deux années de crise sanitaire et de forte inflation, la vie festivalière sera totalement bouleversée, reprogrammée dans les « trous » laissés disponibles par les Jeux, parfois en dehors des vacances scolaires. Dans ce contexte, la politique culturelle du pays se transforme en une gestion de crise et il est difficile de prendre de la hauteur pour adapter nos outils aux grandes transformations en cours.

Après les menaces pesant sur des lieux culturels locaux emblématiques comme Montévidéo à Marseille, on apprend que le prix des loyers chasse les cinémas des Champs Élysées et des cœurs de ville. Il importe donc de les mettre à l’abri de la flambée immobilière, conformément à l’esprit de l’ordonnance de 1945 relative aux spectacles. À nous de nous saisir de la question transversale du partage de la valeur ajoutée dans le secteur culturel et de revaloriser la part des auteurs et des artistes. Les négociations sur les conséquences de l’intelligence artificielle qui ont lieu de l’autre côté de l’Atlantique devraient nous inciter à faire de même, sans plus attendre.

». Comme les formes d’expression pour le dire sont multiples et diverses, qu’elles traversent les âges, les frontières, les ethnies et les religions, la culture est œuvre de communion universelle et intemporelle entre les êtres humains. l’œuvre des politiques publiques devrait être de permettre à chacune et à chacun de s’inviter à cette table de la communion universelle. De ce point de vue, il est positif que les équipements d’enseignement supérieur d’art aient bénéficié d’une aide exceptionnelle de 2 millions d’euros en 2023 pour faire face à la crise et que cette dotation soit pérennisée pour 2024,

afin de permettre à chacune et à chacun de s’instruire, avec plaisir, à partir de la diversité des créations et des productions et – pourquoi pas ? – d’en devenir soi même un acteur. Cela appelle à encourager et à garantir une diversification des politiques de sensibilisation en direction des jeunes. Une approche éducative artistique et culturelle me paraît donc indispensable si nous ne voulons pas que le pass Culture,

pour, finalement, ne pas s’y rendre. Bref, des progrès restent à accomplir pour que ce dispositif, qui demeure un simple outil de politique culturelle, puisse atteindre ses objectifs en matière de démocratisation culturelle. Les crédits du ministère de la culture affichent une hausse de 6 %. Aux côtés de la transition écologique, la lecture, le patrimoine local et la diffusion artistique paraissent en constituer les priorités. La crise sanitaire a durablement affaibli le secteur,

ce sont elles qui fournissent la majeure partie des subventions et des fonds permettant le développement d’une offre de culture variée dans les territoires. Or, nous le savons, elles connaissent toutes une situation de tension

territoriales – en moyenne quatre fois plus que par l’État –, leurs subventions stagnent ou baissent, soit parce que les collectivités sont elles mêmes en difficulté, soit pour des raisons politiques.

c’est une bonne chose. Néanmoins, la restauration du patrimoine de ces communes, notamment du patrimoine religieux, nécessitera un engagement budgétaire spécifique – nous le disons en souhaitant, bien entendu, que les dispositions spécifiques annoncées par le Président de la République trouvent leur pleine efficience. Enfin, je pointerai un un léger regret, celui de l’absence de référence au nécessaire effort à produire pour défendre nos langues et cultures régionales ou minoritaires. La mondialisation et l’uniformisation des standards culturels n’aident pas à la préservation de nos langues. Les locuteurs sont de moins en moins nombreux, aussi peut on craindre une éradication de ces langues, qui participent pourtant de la diversité culturelle du pays. Qu’il me soit permis d’avoir ici une pensée toute particulière pour Édouard Glissant et Eugène Guillevic

Cette année ne fait pas exception et nous le saluons. Toutefois, ce budget présente quelques lacunes que nous souhaitons également souligner, car force est de constater que nombre d’acteurs du secteur sont inquiets.

Ce rééquilibrage doit toucher plusieurs secteurs, en particulier ceux qui se remettent difficilement des années covid. Il appelle à une plus grande concertation entre les acteurs. Ce développement de l’offre doit aussi s’accompagner d’un accès à la culture socialement plus équitable. L’égalité d’accès au savoir culturel est un impératif constitutionnel. Il nous semble essentiel d’accompagner l’augmentation des crédits alloués au pass Culture par des initiatives culturelles tangibles, en garantissant des avantages à l’ensemble de la population, sans favoriser exclusivement les offres des grandes entités industrielles, ce que nous risquons de provoquer si nous n’adaptons pas les politiques dites du chéquier. Les contraintes budgétaires qui pèsent sur les collectivités locales risquent de mettre en péril le spectacle vivant. En effet, leurs marges de manœuvre se réduisent sous l’effet du tassement des ressources et de l’augmentation des charges liées à l’inflation. En conséquence, 30 % de nos collectivités envisagent de réduire leur budget consacré aux projets culturels. Dès lors, une question s’impose à tous : que prévoit le projet de loi de finances pour soutenir la représentation artistique ? Nous saluons les 10 millions d’euros destinés au plan Mieux produire, mieux diffuser, mais nous souhaitons que ces nouveaux crédits puissent justement soutenir les équipements artistiques. les représentants du secteur estiment le besoin des Smac,, à 4 millions d’euros. Que comptez vous faire, madame la ministre ? La situation économique actuelle ne devrait, en aucun cas, justifier des réductions budgétaires dans le domaine des subventions artistiques.

La hausse de la trajectoire des emplois, pour la période allant de 2024 à 2027, est un signal encourageant, afin de conduire une politique que nous espérons encore plus ambitieuse.

Par conséquent, il semble nécessaire de concentrer davantage les moyens de l’éducation artistique et culturelle sur les écoles primaires et maternelles. Il est indispensable que la jeunesse soit sensibilisée, très tôt, à la culture, dans toute sa diversité, qu’elle en soit plus largement à la fois l’actrice et la bénéficiaire, pour son propre épanouissement et dans l’intérêt de la cohésion sociale. L’examen des crédits de cette mission me permet de souligner l’importance de mettre l’accent sur les conditions de circulation de l’information, sur son utilisation et sa véracité. pour nombre de jeunes, hélas !, la culture se concentre dans leur seul téléphone. À l’heure où les plateformes de médias sociaux prennent le relais des médias traditionnels,

Face à ce défi, il devient impératif de mettre en place un plan d’action pour éveiller l’esprit critique de nos jeunes. Cette initiative représente un investissement essentiel pour leur permettre de naviguer, de manière informée et résiliente, au sein d’un environnement complexe et parfois très trompeur.

ces crédits, d’un montant total de 4,2 milliards d’euros en autorisations d’engagement et de 3,9 milliards d’euros en crédits de paiement, sont le reflet d’une politique culturelle ambitieuse, le reflet d’un engagement résolu du Gouvernement en faveur de ce secteur. En effet, la mission « Culture » voit ses crédits augmenter de manière significative, avec une hausse de 11,88 % en autorisations d’engagement et de 4,9 % en crédits de paiement par rapport à l’exercice précédent. Une part prépondérante de cette augmentation est destinée au programme 175 « Patrimoines », avec une progression impressionnante de 32,79 %. Cette impulsion budgétaire s’inscrit dans une politique d’investissement soutenue, mettant en avant des actions cruciales comme la préservation du patrimoine des musées de France, en hausse de 69,06 %, et du patrimoine archivistique, en Ces investissements incluent des projets majeurs, tels que le déménagement des Archives nationales à Pierrefitte sur Seine, la rénovation du centre Pompidou ou encore la création du futur musée mémorial du terrorisme.

de 1,48 milliard d’euros en autorisations d’engagement et de 1,19 milliard d’euros en crédits de paiement, finance la préservation et l’enrichissement du patrimoine culturel français. Le Gouvernement s’engage à valoriser les territoires au travers de leur patrimoine, à soutenir la politique d’archéologie préventive et à investir dans des projets structurants comme la rénovation du grand cloître de l’abbaye de Clairvaux, ancienne abbaye cistercienne et ancienne prison.

culturels. Le programme 361 « Transmission des savoirs et démocratisation de la culture », quant à lui, est doté de 833,3 millions d’euros en autorisation d’engagement et de 828,1 millions d’euros en crédits de paiement. comprend des politiques transversales, allant de l’éducation artistique à la promotion de la langue française. Avec cette dotation, le Gouvernement entend non seulement renforcer les moyens alloués aux écoles de l’enseignement supérieur, tant nationales que territoriales, notamment aux écoles nationales supérieures d’architecture, mais aussi soutenir le pass Culture et mettre en place une stratégie du livre et de la lecture dans les territoires.

Enfin, le programme 224 « Soutien aux politiques du ministère de la culture » est doté de 846,2 millions d’euros en autorisations d’engagement et de 844,3 millions en crédits de paiement. Ce programme soutient la politique internationale et contribue aux fonctions supports du ministère. nous intensifions l’action en matière de politique culturelle internationale, favorisons la transformation numérique et revalorisons les agents du ministère. Examinés de manière approfondie par l’Assemblée nationale, ces budgets ont reçu l’avis favorable de la commission des finances, de l’économie générale et du contrôle

En votant en faveur de ces budgets, nous contribuerons à façonner un avenir culturel riche, diversifié et accessible à tous les citoyens.

Animés par la passion commune de la culture, véritable lien social fédérateur et émancipateur et secteur créateur d’emplois, les acteurs culturels ont besoin d’être soutenus et revalorisés.

Déjà fragilisés par la hausse globale des coûts, ils pourraient avoir à supporter, en 2024, des frais supplémentaires de sécurité, liés à la tenue des jeux Olympiques et Paralympiques. Madame la ministre, vous

de la lecture ou encore de l’éducation aux médias, qui est une priorité impérative à l’heure où se propagent les. Le pass Culture, sévèrement évalué par la Cour des comptes, est seulement un outil

cet engagement est ponctuel et ne règle en rien les questions de fond, qu’elles soient de gouvernance, de statut, d’égalité de traitement des enseignants ou qu’elles concernent les élèves boursiers. Ces questions, que nous avons encore abordées cette semaine avec les commissaires à la culture, trouveront réponse non pas dans le, mais dans des modifications législatives et réglementaires. Enfin, comment ne pas évoquer la place des collectivités territoriales en matière de politiques culturelles ? Or les baisses des dotations de l’État aux collectivités territoriales fragilisent les politiques de proximité, ainsi que le maillage incroyable qui fait notre force collective. Alors que les censures et les entraves à nos libertés fondamentales de création, d’expression et de diffusion ne cessent de croître, nous devons plus que jamais défendre la culture et réaffirmer sa place centrale dans notre société.

Nous devons continuer de défendre la culture comme force émancipatrice, défendre ces actrices et ces acteurs essentiels à notre société. Ce budget doit nous le permettre, très concrètement. Les sénateurs et les sénatrices socialistes voteront ce budget et les amendements présentés par notre collègue Karine Daniel,

L’année 2024 verra la réouverture au public de la cathédrale. La sauvegarde de Notre Dame de Paris est désormais assurée, mais il reste un point d’achoppement : le sort à réserver au surplus de dons, qui dépasse 140 millions d’euros. Le ministère de la culture suggère d’affecter ces fonds au financement de la prolongation de l’établissement public créé et au déploiement d’une troisième phase de travaux. les donateurs étaient pour la plupart animés par la volonté explicite de concourir à l’effort national de reconstruction de Notre Dame. Les deux premières phases de travaux, financées par les fonds récoltés, répondaient en tout point à cette logique. À l’inverse,

l’entretien de tels monuments relève de la responsabilité de l’État. Il ne saurait dépendre de généreux donateurs contribuant par le biais d’une souscription nationale. C’est le moment, me semble t il, d’envoyer un message fort aux acteurs locaux qui se démènent pour tenter de sauvegarder notre patrimoine collectif. Aussi, je vous propose une régionalisation partielle, mais significative de ce surplus, grâce auquel les Drac pourraient concourir à la rénovation de patrimoines religieux très remarquables dans tous les territoires, au lieu de les cantonner à quelques grands projets.

ces écoles ne parviennent plus à équilibrer leur budget ; elles épuisent peu à peu leur fonds de roulement. La reconduction de l’aide d’urgence de 2 millions d’euros accordée en 2023 reste insuffisante, d’où l’amendement de notre collègue Karine Daniel adopté en commission.

la proposition de loi de nos collègues Catherine Morin Desailly, Max Brisson et Pierre Ouzoulias créant un cadre et des mécanismes de contrôle pour ces décisions de restitution.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l’écrivain britannique John Ruskin déclarait à ses contemporains : « Le principe des temps modernes consiste d’abord à négliger les édifices, puis à les restaurer. Prenez soin de vos monuments et vous n’aurez nul besoin de les restaurer. »

outre, depuis l’exercice budgétaire 2023, nous ne pouvons plus compter sur les crédits du plan de relance. Ce budget s’inscrit par ailleurs dans un contexte toujours marqué par la flambée des prix de l’énergie, qui continue de peser fortement sur l’équilibre financier de structures comme les musées et les monuments.

Je pense à la hausse des crédits alloués à l’entretien et à la restauration des monuments historiques, hors grands projets, au fonds incitatif pour le patrimoine ou encore aux études et travaux dédiés aux sites patrimoniaux remarquables.

Plus largement, les carences des moyens humains des services déconcentrés de l’État appellent toute notre vigilance. Il est important de le rappeler : ce sont d’abord nos petites collectivités territoriales qui pâtissent du manque d’agents qualifiés chargés d’accompagner ces projets. ce qui concerne les crédits alloués au patrimoine archéologique, il faut s’interroger sur l’allocation des moyens dégagés par la taxe d’archéologie préventive (TAP), à l’heure où les services territoriaux d’archéologie préventive

En résumé, si nous portons un regard globalement positif sur ce budget en matière de valorisation et de protection du patrimoine, nous émettons quelques réserves quant à sa capacité à répondre à l’ensemble des enjeux auxquels le secteur est confronté.

la culture continue de nous rassembler. Plus que jamais, elle doit nous rassembler. Que ce soit dans l’intimité d’une lecture, dans la moiteur d’une salle de concert – une Smac, peut être ? – ou sous les voûtes majestueuses d’un monument, la culture nous offre des émotions uniques et des imaginaires communs. Elle est le premier chemin vers l’altérité, la compréhension de l’autre, la tolérance et la lutte contre les préjugés. Comment combattre la haine sans la culture ?

de soutenir de nouvelles initiatives, comme la stratégie nationale en faveur des métiers d’art, le fonds d’innovation territoriale ou l’olympiade culturelle. Bien entendu, le budget pour 2024 prend en compte l’inflation, en se fondant sur l’estimation de la Banque de France, à savoir une

pour des appels à projets Alternatives vertes. J’ai également obtenu sur les fonds verts interministériels une enveloppe de 40 millions d’euros pour financer des travaux d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments culturels.

de sujets. En conclusion, j’insiste sur l’importance de notre coopération internationale. Le ministère de la culture travaille main dans la main avec le Quai d’Orsay pour porter la voix de la France dans le monde et tisser de nouveaux partenariats internationaux.

influence dans le monde. « », lit on dans cet article. Oui, nous restons une grande puissance culturelle, une « puissance d’imaginaire », comme disait Malraux. Ce budget historique permet de maintenir et d’amplifier notre ambition.

partout, auprès de l’ensemble des élèves et dans toutes ses composantes.

que de donner à tous les élèves les moyens d’accéder à la culture ? Le pass Culture est un outil pertinent pour y parvenir. Pourquoi ne pas le rendre le plus efficient possible ? Nos communes font d’ailleurs face à une forte demande dans ce domaine de la part des écoles, notamment dans les zones rurales, où il ne suffit pas toujours de traverser la rue